La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 12 décembre 2019 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté. Mes chers collègues, j'ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Jean-Claude Carle, qui fut sénateur de la Haute-Savoie de 1995 à 2018.

les autorités israéliennes viennent d'interdire l'entrée de Jérusalem et de Bethléem aux chrétiens de Gaza. Et alors que des colloques sont organisés de-ci de-là sur la protection des chrétiens d'Orient,

L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi organique et du projet de loi relatifs à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution et prorogeant le mandat des membres de la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet Il a été décidé que ces deux textes feraient l'objet d'une discussion générale commune. Dans la discussion générale commune, la parole est à M. le secrétaire d'État. Monsieur

sénateurs, je suis heureux d'être aujourd'hui devant vous pour vous présenter le projet de loi organique et le projet de loi modifiant les lois organique et ordinaire relatives à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. Le projet de loi ordinaire proroge en outre le mandat des membres de la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi). Il s'agit, pour l'essentiel, de tirer les conséquences de diverses dispositions législatives adoptées récemment, afin de permettre au Parlement de continuer d'exercer son contrôle sur le pouvoir de nomination du Président de la République prévu à l'article 13, alinéa 5, de la Constitution. En effet, en vertu de cet article, le Président de la République nomme « aux emplois civils et militaires de l'État La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a complété cet article d'un cinquième alinéa renvoyant au législateur organique la détermination des « emplois ou fonctions [ ...] pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée ». Ce droit de veto sur certaines nominations décidées par le chef de l'État est une avancée démocratique majeure, pour laquelle il faut rendre hommage au Constituant de 2008 et au législateur organique de 2010. Il est désormais bien ancré dans notre V République que les nominations par décret du Président de la République à des emplois se caractérisant par leur importance, soit pour la garantie des droits et libertés, soit pour la vie économique et sociale, doivent faire l'objet d'un avis préalable des commissions permanentes compétentes des deux assemblées parlementaires. Cette nomination ne peut se faire que lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. Au fil du temps, le législateur organique a eu à compléter la liste prévue par l'article 13, alinéa 5, de la Constitution. Aujourd'hui, ce sont 52 autorités administratives indépendantes (AAI), établissements publics ou entreprises publiques dont les principaux responsables font désormais l'objet d'un tel contrôle parlementaire. Loin d'être une formalité, ces auditions sont un temps politique et, même si le droit de veto n'a jamais encore été mis en oeuvre, elles sont l'occasion pour les commissions d'examiner les compétences des personnes proposées. Ces auditions sont publiques et font l'objet d'un avis public : elles permettent de lancer le mandat de la personne désignée, de lui donner un élan particulier avec une légitimité particulière. Des réformes importantes adoptées ces derniers mois requièrent d'actualiser les lois organique et ordinaire de 2010. Les textes que le Gouvernement vous a présentés, mesdames, messieurs les sénateurs, tirent la conséquence de la loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, qui transforme au 1 janvier 2020 le groupe public ferroviaire constitué de trois établissements publics industriels et commerciaux, en groupe public unifié composé de la société nationale SNCF et de ses filiales directes et indirectes, notamment SNCF Voyageurs et SNCF Réseau. À ce propos, des désaccords subsistent encore sur la gouvernance de l'ensemble, comment ont semblé le montrer Vous le savez, l'ambition de la loi Nouveau pacte ferroviaire était de normaliser la gouvernance du groupe SNCF. Elle le fait, notamment, en ne prévoyant aucune disposition, dans la loi elle-même ou dans l'ordonnance prise sur son fondement, qui fige le cumul ou la dissociation des fonctions de président et de directeur général pour la SNCF ou pour SNCF Réseau.

des lois du Sénat sont probablement motivés par la volonté de garantir l'indépendance du gestionnaire d'infrastructure. Certes, nous partageons cette volonté, mais l'ordonnance prise sur le fondement de la loi Nouveau pacte ferroviaire répond déjà à ces inquiétudes, en prévoyant que la nomination,

L'argent issu de cette privatisation servira à alimenter le fonds pour l'innovation et l'industrie, qui investira dans la durée dans des technologies de rupture, comme l'intelligence artificielle ou la nanoélectronique. Ces textes tirent également la conséquence de l'ordonnance du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard, qui met en place une nouvelle autorité administrative indépendante de régulation du secteur des jeux, l'Autorité nationale des jeux (ANJ). Celle-ci reprend l'intégralité des missions de l'ancienne Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL), en étendant son domaine de compétence à l'ensemble du secteur des jeux d'argent et de hasard, à l'exception des casinos. textes tirent aussi la conséquence de l'ordonnance du 24 juillet 2019 relative au régulateur des redevances aéroportuaires, qui remplace l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (Arafer) par l'Autorité de régulation des transports

de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), aux compétences plus étendues. Les textes dont nous discutons sont essentiellement techniques, de conséquence juridique et d'application pratique. Je note avec plaisir que la commission des lois du Sénat a approuvé les dispositions des projets de loi initiaux. Elle les a même enrichis, soucieuse de bonne légistique et de cohérence juridique. Elle a aussi fait preuve d'une certaine constance dans ses convictions, aux documents administratifs (CADA) à la liste prévue dans la loi organique de 2010. À notre sens, cet ajout n'est pas justifié, la CADA ne satisfaisant pas au critère de « l'importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation », du fait de son rôle presque exclusivement consultatif. De même, l'ajout du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne nous paraît pas opportun, cet organisme ayant également un rôle consultatif important. Le Gouvernement est en revanche pleinement favorable aux autres amendements adoptés par la commission

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la commission des lois a examiné ce projet de loi organique et ce projet de loi ordinaire le 11 décembre dernier. Ils abordent deux sujets distincts : le mandat des membres de la Hadopi et le contrôle, par les commissions parlementaires, des nominations du Président de la République. Initialement, le Gouvernement présentait ces textes comme un travail d'actualisation, voire de coordination. Le diable se cache toutefois dans les détails, et la commission des lois a adopté treize amendements, afin de corriger certaines maladresses. Elle a surtout rappelé son attachement au contrôle parlementaire sur les nominations aux emplois publics.

Il ne veut pas nommer de nouveaux membres, alors que la Haute Autorité devrait fusionner avec le CSA le 25 janvier 2021. Le Gouvernement souhaite également que l'actuel président de la Hadopi continue son travail de préfiguration, pour bien préparer cette fusion. La commission des lois ne s'est pas opposée à cette disposition, dont la portée reste limitée. L'examen de l'amendement de notre collègue David Assouline permettra d'en débattre de manière plus approfondie. J'en viens à la procédure prévue au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. Créée par la révision constitutionnelle de 2008, elle permet au Parlement de bloquer une nomination du Président de la République lorsque l'addition des votes négatifs dans les commissions compétentes représente, au total, au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés c'est ce que l'on appelle parfois les « trois cinquièmes négatifs ». Cette procédure concerne aujourd'hui 54 emplois, qui présentent une « importance particulière pour les droits et libertés ou pour la vie économique et sociale de la Nation

Depuis 2011, le Parlement s'est exprimé à 110 reprises sur des nominations envisagées par le Président de la République. Il n'a jamais mis en oeuvre son pouvoir de veto, ce qui a d'ailleurs conduit le groupe de travail du Sénat sur la révision constitutionnelle à proposer une modification des règles de blocage. À six reprises, l'une des commissions compétentes a formulé un avis négatif, marquant son désaccord sur le projet de nomination. Je rappelle notamment l'opposition du Sénat à la nomination d'un membre du Conseil supérieur de la magistrature, le CSM, qui souhaitait, à titre temporaire, cumuler cette fonction avec celle d'ambassadeur de France à Madrid ... La plupart d'entre nous s'en souviennent, c'est assez récent. Le dernier exemple date de la semaine dernière. La commission des affaires économiques du Sénat s'est opposée à la nomination du directeur général de l'Office national des forêts. Il s'en est fallu d'une seule voix pour bloquer la nomination Avec ces projets de loi, le Gouvernement propose d'actualiser la liste des nominations soumises à l'avis préalable des commissions parlementaires. Certaines dispositions ne soulèvent aucune difficulté,

Le Gouvernement propose également de supprimer le poste de P-DG de la Française des jeux de la liste de l'article 13 de la Constitution. Nous gardons tous en mémoire l'opposition qu'a exprimée le Sénat sur le projet de privatisation de la société.

les textes du Gouvernement soulèvent un problème de méthode et un problème de fond, qui dépassent un simple exercice de toilettage. Sur le plan de la méthode, nous sommes invités à tirer les conséquences de trois ordonnances qui n'ont pas encore été ratifiées, sur des sujets aussi importants que la police des jeux ou l'organisation du réseau de transport. Alors qu'elle réorganise entièrement la SNCF, l'ordonnance du 3 juin 2019 n'a toujours pas été ratifiée, plus de six mois après sa publication.

Sur le fond, les projets de loi initiaux conduisaient à un recul, même léger, du contrôle parlementaire sur les nominations aux emplois publics. La commission des lois n'a pas accepté cette évolution, qui serait allée à rebours des efforts accomplis depuis 2009 pour renforcer cette procédure de contrôle et élargir son périmètre.

Pour la première fois depuis 2010, le Parlement aurait perdu tout droit de regard sur la gouvernance du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, SNCF Réseau, ce qui n'était pas acceptable. SNCF Réseau doit, au contraire, bénéficier de garanties d'indépendance suffisantes, pour éviter toute discrimination entre les entreprises de transport, dont SNCF Voyageurs. En conséquence, le texte de la commission soumet au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution le président du conseil d'administration et le directeur général de la société nationale SNCF, mais également celui de SNCF Réseau. Dans la même logique, la commission des lois a ajouté deux fonctions à la liste des nominations soumises à l'avis préalable des commissions parlementaires : le président de la Commission d'accès aux documents administratifs et le et le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Nous avons travaillé de conserve avec Jean-Yves Leconte pour obtenir ce résultat, qui me semble très satisfaisant. La mission de en matière d'accueil des demandeurs d'asile et des immigrés s'est fortement affirmée au cours des dernières années. Pour la seule année 2018, l'OFII a organisé le premier accueil de 109 783 demandeurs d'asile. Il a également conclu 97 940 contrats d'intégration républicaine, qui permettent aux étrangers d'accéder à des formations linguistiques, donc de mieux s'intégrer à la société française.

numérique a même étendu ses missions, lesquelles couvrent désormais la publication en open data des documents administratifs et la réutilisation d'informations publiques.

Nous souhaitons donc vous interpeller, monsieur le secrétaire d'État, sur la situation de cette autorité administrative indépendante, qui n'arrive plus à faire face au volume et à la complexité des demandes reçues. En 2018, la CADA a été saisie de 5 867 demandes d'avis. En moyenne, chaque dossier a été traité en 128 jours, alors que la loi fixe un délai théorique de 30 jours. Une fois la décision de la CADA rendue, les citoyens doivent encore attendre deux mois pour obtenir une réponse de l'administration et, le cas échéant, pour se porter devant le tribunal administratif. C'est un véritable labyrinthe ! En commission, nombre de collègues ont également mentionné les élus d'opposition, qui, dans leurs assemblées, ne parviennent dans leurs assemblées, ne parviennent pas à obtenir des documents dans les temps. De l'aveu même de son président, la CADA ne peut plus continuer ainsi. Son « stock d'affaires » s'élève actuellement à 1 800 dossiers, ce qui correspond à environ quatre mois d'activité. Quelles solutions envisagez-vous, monsieur le secrétaire d'État, pour mettre fin à cette situation, alors que les citoyens sollicitent de plus en plus l'accès aux documents administratifs ? Il s'agit, vous l'aurez compris, d'un sujet essentiel pour le Sénat. Plus globalement, nous regrettons l'attitude du Gouvernement qui a déposé tardivement sept amendements visant à revenir sur les amendements de la commission

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la réforme ferroviaire, que nous avons adoptée il y a près d'un an et demi, prévoit une évolution profonde de la gouvernance de la SNCF, qui passera au 1 janvier 2020 du statut de groupe public ferroviaire constitué d'EPIC à celui de groupe public unifié constitué de sociétés anonymes. Cette évolution doit être précisée par ordonnance. Or cette ordonnance, publiée au mois de juin dernier, n'a pas été ratifiée par le Parlement, et aucun calendrier de ratification ne m'a été communiqué. d'État, pourriez-vous nous en dire plus sur le calendrier de ratification envisagé ? En outre, l'Autorité de régulation des transports a émis de sérieuses réserves sur son contenu, en particulier sur l'indépendance du gestionnaire d'infrastructure, SNCF Réseau. Réseau. Elle a d'ailleurs réitéré ses craintes dans son récent avis sur les projets de décrets statutaires des sociétés du futur groupe public unifié. Les projets de loi organique et ordinaire que nous examinons aujourd'hui entendent pourtant tirer les conséquences des dispositions de cette ordonnance. Au-delà de cette méthode, que je qualifierais de discutable, ces textes conduiraient à affaiblir le contrôle parlementaire sur la nomination des dirigeants de la SNCF, puisqu'ils prévoient de remplacer les trois auditions actuellement prévues par une unique audition du directeur général de la société nationale SNCF maison mère. Or l'évolution de la gouvernance du groupe ne saurait justifier de restreindre ainsi le droit de regard du Parlement sur de telles nominations. La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable s'est saisie pour avis de ce texte et a entendu, avec l'avis favorable de la commission des lois, conforter le contrôle parlementaire sur la nomination des dirigeants de la SNCF, selon trois axes. Tout d'abord, la commission a veillé à maintenir la procédure prévue à l'article 13 de la Constitution pour la nomination du dirigeant de SNCF Réseau, qui est prévue depuis 2010 et que le projet de loi organique tendait pourtant à supprimer. Or avoir choisi de maintenir une structure verticalement intégrée justifie à plus forte raison d'encadrer la nomination du dirigeant de la société SNCF Réseau. Aussi, en raison du rôle central que jouera le gestionnaire d'infrastructure dans l'accès au réseau et dans la perspective de l'ouverture à la concurrence, la commission a-t-elle été soucieuse de garantir l'audition de son directeur général par les commissions compétentes du Parlement. Ensuite, étant donné que la possibilité sera laissée au conseil d'administration de la société mère et de la filiale SNCF Réseau de dissocier la direction générale de la présidence du conseil d'administration et en raison du rôle important que jouera le président du conseil d'administration dans chacune de ces sociétés,

déposé par les députés dans le cadre de l'examen du projet de loi portant réforme ferroviaire de 2014. En effet, ils sont toujours d'actualité : « Il est impératif que les processus de nomination des dirigeants du futur groupe public ferroviaire continuent de se dérouler sous le regard des parlementaires. Nul ne comprendrait ni n'admettrait que la réforme soit l'occasion de soustraire ces personnalités à un contrôle qui constitue une avancée unanimement reconnue de la démocratie. » Enfin, un amendement au projet de loi ordinaire vise à soumettre la nomination du président du conseil d'administration de la société SNCF Réseau à l'avis conforme de l'ART, alors que l'ordonnance ne réserve cette procédure qu'au directeur général ou, le cas échéant, au président-directeur général. Les choix en matière de gouvernance et les modalités de nomination des dirigeants du groupe contribuent en effet à garantir cette indépendance. Aussi, dans le contexte de l'ouverture à la concurrence du transport national de voyageurs et alors même que le régulateur et les nouveaux entrants ont exprimé de vives inquiétudes, il est essentiel de veiller à garantir les conditions d'indépendance du gestionnaire d'infrastructure. En conclusion, les amendements adoptés par la commission des lois, sur proposition de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, visent à renforcer le contrôle du Parlement

nous sommes appelés aujourd'hui à légiférer sur un double sujet : d'une part, l'actualisation de la liste des nominations du Président de la République soumises à l'avis préalable des commissions parlementaires, conformément à la procédure dite « des trois cinquièmes négatifs », ce qui représente 54 emplois aujourd'hui

que la prolongation des mandats des membres de la Hadopi concernerait les membres titulaires, mais également leurs suppléants. Elle a également pris acte du changement de nom de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la Banque publique d'investissement, La commission des lois a également souhaité intégrer le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ainsi que le président de la Commission d'accès aux documents administratifs à la liste des emplois concernés par cette procédure de contrôle. Nous n'avons aucun préjugé défavorable quant au nombre de désignations devant être opportunément soumises au contrôle du Parlement. Encore faut-il que l'OFII, en sa qualité d'organisme consultatif, s'inscrive, en droit, dans le champ de l'article 13 de la Constitution, ce dont nous pouvons légitimement douter. Par ailleurs, l'effervescence suscitée par les modalités de nomination des dirigeants de la société nationale SNCF et de SNCF Réseau semble inversement proportionnelle à l'intérêt de cette affaire. En effet, en l'état, le régime commun des sociétés à participation publique prévoit que que seul le mandataire social d'une société directement détenue à plus de 50 % par l'État est nommé par un décret du Président de la République. Nous sommes également dubitatifs s'agissant de la réaction de principe consistant à dire que ce véhicule législatif préjugerait, en toute hypothèse, de processus de ratification ultérieurs : si nous en comprenons la rentabilité politique, la logique juridique semble nous échapper. Politiquement, il peut être en effet avantageux de soupçonner autre chose qu'un texte de coordination. Juridiquement, en revanche, c'est sans doute un peu cavalier : les ordonnances, quoiqu'elles soient dépourvues de valeur législative, produisent d'ores et déjà leurs effets administratifs et sollicitent, par ce fait même, un certain nombre de coordinations. Il ne faut donc y voir aucun blanc-seing ou négation du contrôle parlementaire. Au reste, les dispositions présentées dans ces projets de loi restent circonscrites à un champ normatif très limité et n'appellent pas d'observation particulière de notre part, exception faite, peut-être, de notre souhait de voir figurer, en bonne place, une réelle rationalisation de cette nébuleuse infiniment complexe que sont les autorités administratives indépendantes.

La version finale de l'article 13 est bien différente, il faut le rappeler, afin de bien mettre en évidence le contresens démocratique : « Le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. » À ce stade, il ne s'agit que d'un simple avis, nullement impératif. L'article prévoit ensuite : « Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions ».

Un véritable pouvoir de contrôle, assorti de moyens d'influer sur la réalité et d'une véritable transparence, est devenu un impératif démocratique, tant la critique contre les institutions devient forte, comme nous pouvons le noter à l'occasion de la désastreuse affaire Delevoye. Comment ne pas faire le lien entre ces remarques et la légèreté, pour ne pas dire le peu de respect, qui conduit le Gouvernement à proposer d'adapter la liste prévue par la loi organique, afin de prendre en compte la nouvelle gouvernance de la SNCF à la suite de la modification de ses statuts ?

Les dispositions relatives à la nouvelle gouvernance du groupe ont été précisées dans une ordonnance de juin 2019, qui n'a pas été ratifiée par le Parlement et qui fait par ailleurs l'objet de nombreuses réserves. Je constate donc qu'il nous est aujourd'hui demandé de nous prononcer sur des textes entérinant des choix sur lesquels nous n'avons pas eu l'occasion de débattre ». Si cette remarque est judicieuse, je rappellerai néanmoins que nous sommes bien souvent seuls sur les travées du groupe CRCE à contester la multiplication du recours à la pratique des ordonnances ! Je partage le souhait des deux commissions d'adapter le contrôle de la gouvernance de la SNCF. Je m'interroge toutefois sur vos motivations profondes, mes chers collègues, car l'un de vos premiers soucis semble être d'écarter toute gêne dans la mise en oeuvre de la politique d'ouverture

Ces projets de loi organique et ordinaire sont donc loin d'être anecdotiques. Ils sont dans l'air du temps- un air assez mauvais. L'heure est à la mise à l'écart du Parlement, à une présidence de la République toute-puissante, à un marché profitant à plein régime de ces défaillances démocratiques.

soumises à l'avis préalable des commissions parlementaires et à prolonger le mandat de six membres de la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet. Depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la V République, le Parlement dispose d'un pouvoir de veto sur certaines nominations effectuées par le Président de la République en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation », comme le prévoit le cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. Ces nominations sont soumises à l'avis préalable des commissions compétentes de chaque assemblée. Le Président de la République doit y renoncer lorsque l'addition des votes négatifs représente, au total, au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés. Cette procédure de contrôle repose sur deux piliers juridiques : la loi organique du 23 juillet 2010, qui dresse la liste des 54 emplois concernés, et la loi ordinaire de la même date, qui précise la procédure applicable, ainsi que les commissions compétentes. Un tel contrôle parlementaire apparaît indispensable. En effet, l'avis préalable des commissions parlementaires présente un double intérêt. D'une part, il renforce le contrôle des nominations par le Président de la République d'autre part, il garantit la transparence de ces nominations, notamment grâce à l'audition des candidats pressentis. Si la liste des emplois relevant du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution a été modifiée à treize reprises depuis 2009, elle n'a toutefois jamais fait l'objet d'un toilettage complet de la part du législateur. Le projet de loi organique et le projet de loi ordinaire qui nous sont soumis aujourd'hui visent à actualiser cette liste, notamment pour tirer les conséquences de mesures prises par des ordonnances récentes. Les mandats de six membres de la Hadopi seraient prolongés jusqu'au 25 janvier 2021, dont ceux du président du collège et de la présidente de la commission de protection des droits. Le Gouvernement ne souhaite pas nommer de nouveaux membres d'ici à cette date, alors que le futur projet de loi sur l'audiovisuel devrait prévoir la fusion de la Si le projet de loi organique et le projet de loi ordinaire sont présentés comme des textes de coordination, ils soulèvent toutefois une difficulté de fond, car ils conduisent à un léger recul du contrôle parlementaire sur les nominations

Cette évolution irait à rebours des efforts consentis depuis 2009 pour renforcer cette procédure de contrôle et élargir son périmètre. Dans ce contexte, je me félicite donc que la commission des lois ait consolidé les dispositifs existants. Elle a notamment précisé que la prolongation des mandats des membres de la Hadopi concernerait les membres titulaires, mais également leurs suppléants. Elle a également pris acte du changement de nom de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la Banque publique d'investissement, Bpifrance, que chacun de vous connaît, mes chers collègues. De même, je me félicite de l'initiative de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, qui a prévu de soumettre quatre dirigeants de la SNCF à la procédure prévue au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. Dans le même esprit, je suis heureux que la commission des lois ait souhaité que le Parlement se prononce sur la nomination, par le Président de la République, du président de la commission d'accès aux documents administratifs, ainsi que du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont la mission s'est fortement affirmée au cours des dernières années.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, en 2008, l'introduction d'un cinquième alinéa à l'article 13 de notre Constitution fut l'une des innovations destinées à « reparlementariser » nos institutions, selon l'expression du constitutionnaliste Jean Gicquel. D'inspiration américaine, cette disposition visait à étendre le contrôle des assemblées à certaines nominations au sein de l'administration qui sont effectuées par le Président de la République « en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation Ce contrôle a également été introduit au moment où l'activité administrative se recomposait. C'est en grande partie la conséquence de l'influence du droit de l'Union européenne, qui a entraîné la prolifération d'autorités de régulation du secteur économique, afin de réduire au strict minimum les interférences entre la sphère politique et la sphère économique, dans une stricte logique libérale. Les pouvoirs autrefois dévolus à des services placés sous l'autorité de ministres sont donc à présent confiés à des autorités administratives à géométrie variable, qu'elles prennent la forme d'autorité administrative indépendante ou d'agence. Comme l'avait noté notre ancien collègue Jacques Mézard dans un rapport qui continue de faire référence, leur indépendance à l'égard du politique varie d'une autorité à l'autre, malgré les tentatives de simplification. Dans tous les cas, elle soulève un problème de responsabilité et de faculté à rendre compte de ses actes devant les représentants de la Nation, comme autrefois les ministres sous l'autorité desquels ces actes étaient pris. Dans ce contexte, il était devenu impératif d'associer le Parlement à ces nominations, ainsi qu'à celles aux fonctions de direction des autorités chargées de la défense des droits et libertés de nos concitoyens, afin qu'il puisse jouer son rôle de contre-pouvoir, même. Si

Dans le détail, en effet, les dispositions proposées par le Gouvernement s'inscrivent dans la continuité de récentes réformes de différents secteurs économiques, anticipant même parfois leur entrée en vigueur. Les plus fins juristes de cette assemblée ont déjà évoqué les limites juridiques d'une telle impatience ... Attention à ne pas réduire la ratification d'une ordonnance à une simple formalité ! Je n'y reviendrai pas. Certaines des modifications proposées ont une faible portée et visent parfois à procéder à de simples coordinations. Je pense au remplacement de l'Arafer par la nouvelle Autorité de régulation des transports dans la liste par exemple Comme l'a souligné notre rapporteur, d'autres modifications sont plus problématiques, car elles réduisent le champ du contrôle exercé par le Parlement et s'inscrivent à rebours de l'Histoire. C'est le cas des nominations au sein de la SNCF, à la suite de la transformation du groupe national ferroviaire. Nous accueillons donc avec beaucoup de satisfaction les modifications introduites en commission, lesquelles visent à maintenir un droit de regard minimal des élus de la Nation sur le fonctionnement interne de ces structures d'intérêt national.

tout d'abord déposé un amendement visant à proposer l'intégration de la direction générale de l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information à la liste. L'importance de la mission de cette autorité, tant pour la vie économique de la Nation que pour la garantie des droits et des libertés en ligne de nos concitoyens, ne fait aucun doute.

qui agite les théoriciens du droit, mais qui a également mobilisé le Conseil d'État, lequel a, en 2017, rejeté une requête du président du Sénat tendant à l'annulation d'une nomination. La décision des juges de la place du Palais royal contraint désormais les commissions parlementaires à se prononcer dans un délai raisonnable de huit jours.

Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, et dans la continuité de nos travaux précédents, nous proposons d'aborder ce sujet par la question du contenu du contrôle effectué, en prévoyant notamment, dans le projet de loi organique, que celui-ci a particulièrement pour objet de lutter contre les cumuls et de prévenir les conflits d'intérêts. De façon générale, nous serons particulièrement attentifs à toutes les initiatives destinées à renforcer la qualité de ce contrôle, afin de le rapprocher davantage de celui effectué dans d'autres démocraties, comme les États-Unis. La parole

le contrôle par les chambres du pouvoir de nomination du Président de la République est encore très timide depuis sa création en 2008. Il nous paraît nécessaire de muscler la procédure d'avis devant nos chambres parlementaires, afin de s'assurer de la qualité des candidatures proposées aux fonctions déterminantes pour les droits et libertés de nos concitoyens et pour le bon fonctionnement de notre économie. Il s'agit de garantir que cette confirmation ne soit pas perçue comme une simple formalité par les personnes nommées, au point que certaines démissionnent parfois de leurs précédentes fonctions avant même d'avoir entendu l'avis des parlementaires Les textes sont assez laconiques. L'article 13 de la Constitution édicte seulement les règles de majorité avec une majorité de blocage de trois cinquièmes, ce que nous avons toujours contesté. L'article 5 de l'ordonnance de 1958 prévoit par ailleurs que le scrutin doit être dépouillé simultanément dans les assemblées.

Or, compte tenu de problématiques déjà soulevées à maintes reprises, liées à la mobilité des hauts fonctionnaires, nous souhaiterions pour commencer inscrire dans la loi organique que l'audition conduite dans les chambres

Parmi les failles les plus récentes, on a par exemple pu lire que La Poste avait « laissé 23 millions de données d'entreprises en accès libre », la caisse en ligne Genius. Ce problème touche également les particuliers. Récemment, le géant Samsung avait recommandé aux utilisateurs de certains de ses téléphones de supprimer leurs empreintes digitales. Et Google a révélé que les failles des iPhone de son concurrent Apple permettaient à des hackers d'accéder aux photos, géolocalisations et données de ses utilisateurs. L'État est également concerné, puisque 2 000 comptes fiscaux de contribuables auraient été piratés. La protection des systèmes d'information est donc l'affaire de tous. Elle remplit les deux cas de figure prévus au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. C'est pourquoi nous proposons que le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'Anssi, soit nommé selon ces modalités, afin que les parlementaires puissent s'assurer, avec le Premier ministre

Toutefois, cet amendement nous paraît très fragile sur le plan constitutionnel. En effet, l'Anssi est un service national à compétence nationale rattaché au Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, donc au Premier ministre, responsable de la défense nationale, est chargé de définir la politique gouvernementale en matière de sécurité. Il s'agit donc d'un service administratif, qui n'est pas couvert par le cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. cet amendement soulèvent également un problème de principe. Le Président de la République nommerait un agent directement placé sous la hiérarchie du Premier ministre. Vous voyez que c'est un peu compliqué ... Pour toutes ces raisons, je demande

rattaché à une administration centrale, le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, le SGDSN. Il ne s'agit pas, comme les organismes mentionnés par l'article 13, d'un établissement public, d'une autorité administrative indépendante ou d'une autre personne morale non soumise à l'autorité hiérarchique directe du Gouvernement. Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information à rang de directeur d'administration centrale. Sa nomination relève donc du troisième alinéa de l'article 13 de la Constitution,

le secrétaire d'État. L'emploi de président de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) n'entre pas dans le périmètre de la procédure prévue au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. Son action vise principalement à faciliter l'accès aux documents administratifs. La CADA rend presque exclusivement des avis, qui sont un préalable éventuel à la saisine du juge administratif. Cependant, elle ne dispose pas d'un pouvoir coercitif. Seul le juge administratif est compétent pour enjoindre à l'administration la communication d'un document. Son rôle consultatif, bien qu'incitatif à l'égard de l'administration, est limité dans sa portée. Le pouvoir de sanction dont elle a été récemment investie en cas de violation des règles de réutilisation des informations publiques n'est qu'accessoire à cette activité principale. La cohérence des emplois et fonctions mentionnés par le cinquième alinéa de l'article 13 s'oppose dès lors à ce que le président de la CADA soit intégré à la liste des emplois et fonctions visés par cette procédure. C'est d'ailleurs la position qui a été retenue lors des débats parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes : l'ajout de la présidence de la CADA avait alors été rejeté. À nos yeux, aucune circonstance nouvelle ne justifie de revenir aujourd'hui sur une telle position. Le Gouvernement souhaite donc supprimer le président de la CADA de la liste des autorités soumises à cette procédure.

la CADA, qui joue un rôle majeur dans le droit d'accéder aux documents administratifs. L'argumentaire du Gouvernement relève d'ailleurs d'une interprétation erronée de l'article 13 de la Constitution, qui n'exclut pas les organes consultatifs. Ainsi, la Commission de contrôle du découpage électoral est déjà soumise à cette procédure, alors qu'elle se limite à rendre un avis public ; je renvoie le Gouvernement à l'article 25 de la Constitution.

Il faut revenir au texte même de l'article 13 de la Constitution. La transparence et le contrôle du Parlement sur les nominations du Président de la République concernent notamment les postes ayant une importance particulière pour la garantie des libertés publiques.

Nous avons le sentiment que vous considérez déjà la CADA comme un organe totalement consultatif. C'est très regrettable. Je ne vois pas comment nous, parlementaires, allons pouvoir effectuer notre travail si l'on nous empêche d'accéder aux pièces des administrations.

: « L'État continuera à agréer les dirigeants de l'entreprise ». C'est donc une entreprise privée d'un type particulier. D'ailleurs, vous le savez, la Française des jeux continuera à servir les intérêts de l'État, notamment financiers et fiscaux. En effet, celui-ci conservera l'intégralité des recettes fiscales et sociales versées à la Française des jeux, soit la modique somme de 3,5 milliards d'euros.

est contraire à la Constitution. Depuis son entrée en bourse, la Française des jeux est une entreprise privée. Or l'article 13 de la Constitution concerne uniquement les emplois publics, qu'ils soient civils ou militaires. Juridiquement, la nomination du P-DG d'une telle structure ne peut donc plus relever du Président de la République. Comme je l'ai indiqué dans le rapport,

Il ne fait guère de doute que cet établissement public est un acteur essentiel en matière d'accueil des étrangers et d'asile. Cependant, il ne formule que des avis destinés au préfet et ne se prononce pas sur le droit au séjour en matière d'asile. Il exerce certaines de ses missions dans le cadre défini par le ministère chargé de l'asile ou pour le compte de ce dernier. Son rôle d'appui, de coordination et de consultation ne répond donc pas aux critères définis au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.

Il organise les procédures de regroupement familial et le retour volontaire. Enfin, c'est l'OFII qui organise les visites médicales des étrangers en France, notamment lorsqu'ils demandent un titre de séjour. L'OFII joue donc un rôle majeur, au même titre que l'Office Il garantit les droits des ressortissants étrangers et doit relever à ce titre du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.

de mise en danger de l'indépendance de SNCF Réseau au sein de la SNCF, et il a même considéré que le texte était compatible avec la directive européenne. Par ailleurs, me semble important de ne pas déroger au droit commun des sociétés à participation publique défini par l'ordonnance du 20 août 2014 : seul le dirigeant mandataire social d'une société détenue directement à plus de 50 % par l'État est nommé par décret du Président de la République. Dans la

dans un contexte d'ouverture à la concurrence du secteur ferroviaire, SNCF Réseau doit bénéficier de garanties suffisantes d'indépendance, pour éviter toute discrimination entre les différentes entreprises de transport, dont SNCF Voyageurs. C'est d'ailleurs l'avis du président de l'Autorité de régulation des transports, que j'ai auditionné au début du mois. Contrairement au Gouvernement, nous souhaitons également un contrôle sur la nomination des présidents du conseil d'administration de la SNCF

L'application du droit commun des sociétés à la SNCF doit se faire avec un minimum de discernement. La SNCF et, plus encore, SNCF Réseau ne sont assurément pas des entreprises comme les autres. Alors que l'indépendance de SNCF Réseau est menacée- L'ART l'a rappelé très récemment dans son avis sur les projets de décrets statutaires -, et alors même que nous entrons dans une phase d'ouverture à la concurrence, il est plus que jamais nécessaire de maintenir le droit de regard du Parlement sur ces nominations. Je me permets d'insister, en particulier, sur la nomination du dirigeant du gestionnaire d'infrastructure, SNCF Réseau, pour lequel la procédure s'applique depuis 2010 et a été réaffirmée en 2014.

13 de la Constitution. En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit. Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

Le scrutin est clos. J'invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

Actuellement, l'article 1 de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution prévoit que ces auditions sont publiques, sauf deux hypothèses : la préservation du secret de la défense nationale et la préservation du secret professionnel. Si la Si la première exception est légitime, l'expérience permet aujourd'hui de dire que la seconde n'est pas fondée. Cette restriction nous semble inopportune s'agissant d'une audition visant à évaluer la candidature soumise par le Président de la République à un emploi ou une fonction relevant de l'article 13. En tout

du règlement de l'Assemblée nationale, qui devrait donc être modifié en conséquence. J'appelle donc à la prudence sur ce point, en vous rappelant que toute personne qui rompt ce secret est passible d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, conformément à l'article 226-13

cet amendement, qu'il n'y a pas de droit ou de devoir de réserve, mais seulement une obligation de discrétion professionnelle, qui ne s'applique qu'aux fonctionnaires encore en poste au moment de leur audition et pour les seuls éléments qui concernent l'exercice de leurs fonctions actuelles. Il est vraiment

l'avis du Parlement constitue une garantie d'indépendance pour le candidat pressenti, mais forcer celui-ci à répondre conduirait à une impasse. En effet, soit la réponse du candidat se limitera à une déclaration d'intention, qu'il sera impossible de contrôler, soit soit sa prise de position pourrait être considérée comme un mandat impératif, ce qui ne correspond pas à l'esprit de l'article 13 de la Constitution. Il nous semble donc préférable d'en rester au droit en vigueur. En pratique, chaque parlementaire peut adapter le sens de son vote en fonction des réponses ou de l'absence de réponse des candidats.

commission ? L'Anssi est un service à compétence nationale, rattaché au Premier ministre. Prévoir une nomination par le Président de la République ne me paraît pas constitutionnel. De même, la Constitution ne prévoit pas que les nominations effectuées par le Président de la République lui soient proposées par le Premier ministre.

il est extrêmement désagréable pour le Parlement de tenir pour acquis le vote d'une loi, dont le projet vient seulement d'être adopté en conseil des ministres et dont l'inscription à l'ordre du jour semble devoir être différée.

conduirait à supprimer l'introduction d'un avis conforme du régulateur sur la nomination du président du conseil administration de SNCF Réseau qui existe actuellement. Le choix de maintenir une structure verticalement intégrée justifie à plus forte raison les modalités de nomination de ses dirigeants, et pas uniquement de son directeur général comme le prévoit l'ordonnance. Les modalités de nomination reflètent, au moins en partie, le degré d'indépendance du gestionnaire de réseau

la commission, modifié, le projet de loi modifiant la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution et prorogeant le mandat des membres de la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet. La parole

d'application du droit sur le territoire national et les modalités d'application dans le temps des dispositions envisagées. Autant de points qui seraient

mesdames, messieurs les sénateurs, je suis très heureux d'être devant vous aujourd'hui afin de pouvoir étudier ce texte relatif à la lutte contre la haine en ligne. Rares sont en effet les textes qui répondent à un besoin aussi pressant et à une demande aussi forte de nos concitoyens, celle d'assurer leur sécurité et de faire respecter leurs droits et leurs libertés, en ligne comme hors ligne. Les malheureux événements de Noisiel survenus à la fin du mois de novembre nous l'ont rappelé une énième fois : internet et les réseaux sociaux peuvent être de formidables vecteurs de démocratie et de connaissance- sans eux, pas de révolutions arabes mais ils peuvent aussi être synonymes du pire. Il suffit de passer quelques instants sur Twitter, YouTube ou Facebook pour y croiser menaces de mort, injures homophobes, banalisation du racisme et de l'antisémitisme. La haine a, presque quotidiennement, libre cours sur internet et les premières victimes parmi nos concitoyens sont les plus jeunes, les plus fragiles et les personnes issues de minorités.

douleur est amplifiée par les réseaux sociaux qui diffusent d'autant plus un contenu qu'il fait réagir, quitte à amplifier massivement une humiliation, une diffamation ou des propos chargés de haine. Cette violence, peu à peu, fragilise notre lien social. La douleur des victimes est amplifiée par le sentiment d'impuissance et d'isolement auquel elles sont confrontées : c'est notamment vrai lorsqu'un réseau social laisse beaucoup trop longtemps en ligne l'un de ces contenus ou que leur auteur peut s'abriter derrière une quasi complète impunité de fait, alors même qu'il a proféré une injure ou une menace punie par la loi française.

Lorsqu'une victime doit fuir, s'isoler, s'excuser, lorsque certains se sentent moins légitimes ou intégrés parce qu'ils se font quotidiennement insulter ou menacer en ligne en toute impunité, lorsque ceux qui les agressent se sentent ignorés par les autorités et peuvent agir impunément, alors c'est le douloureux syndrome de notre échec et de notre impuissance et c'est, pour nous tous, mais d'abord pour l'État, une lourde responsabilité. Disons-le encore plus clairement

ce qui se passe sur internet sont des pays autoritaires, alors les citoyens se tourneront vers des solutions autoritaires ! Raisonnement intéressant ! C'est pour répondre à cette urgence que le Président de la République a souhaité confier à la députée Laetitia Avia l'élaboration de cette proposition de loi qui vise à prendre en compte le rôle majeur que les réseaux sociaux jouent désormais dans nos relations sociales et les responsabilités qui leur incombent à ce titre. Ce texte a été longuement mûri, d'abord grâce au rapport produit par Laetitia Avia, Gil Taïeb et Karim Amellal, ensuite dans le cadre de la mission lancée auprès de l'entreprise Facebook pour mieux comprendre le fonctionnement des processus de modération, mais aussi les multiples consultations qui ont eu lieu avec la société civile et avec nos partenaires étrangers.

Le parcours parlementaire de ce texte a permis de préciser les trois objectifs forts qui sont ceux du Gouvernement et qui forment la colonne vertébrale de cette proposition de loi. Tout d'abord, la conviction que c'est bien l'État qui est le premier responsable pour faire respecter les droits et libertés en ligne. C'est pourquoi il est déterminant de mieux outiller les autorités, en particulier les autorités judiciaires, pour lutter contre le sentiment d'impunité qui prévaut actuellement et punir effectivement les auteurs de contenus haineux. C'est pour cela que la garde des sceaux a annoncé la spécialisation d'un parquet sur ces enjeux numériques et le déploiement progressif de dispositifs de plainte en ligne. Le rôle de la justice est bien au coeur de ce texte qui a vocation à le renforcer. Ensuite, une responsabilité particulière des plus grandes plateformes dans la lutte contre les contenus odieux de loi ne fait que renforcer des principes déjà posés depuis la loi pour la confiance dans l'économie numérique, mais elle rend ces obligations opérationnelles, en les précisant et en les accompagnant d'obligations de moyens et d'une véritable supervision qui constituent le coeur et la vraie innovation de ce texte. Enfin, la mobilisation de toutes les parties prenantes est organisée en matière d'éducation et d'information. Évidemment, il s'agit de priorités qui se prêtent moins à l'exercice législatif, mais nous avons la conviction que l'éducation, la sensibilisation des plus jeunes et l'information des victimes comme des auteurs constituent certaines des armes les plus efficaces pour éradiquer durablement la violence en ligne. Cette priorité est déclinée à la fois en matière d'éducation au sens strict, mais aussi la création d'un observatoire de la haine en ligne pour mieux prendre en compte ce phénomène. Bien sûr, nous avons entendu certaines inquiétudes sur l'impact de ce texte, notamment les craintes de sur-censure. Il s'agirait évidemment d'un écueil majeur, qui est au coeur de nos préoccupations depuis le début et contre lequel l'Assemblée nationale a déjà largement renforcé les garde-fous. Entre la protection nécessaire des victimes et le respect vigilant de la liberté d'expression, j'ai parlé à l'Assemblée nationale d'une ligne de crête qu'il nous faut respecter. Tout en soulignant et en saluant le nouveau cadre de régulation créé par la loi, le Sénat s'est inquiété de ce risque de sur-censure et a, conséquemment, apporté un certain nombre de modifications à l'article 1. J'estime que ces modifications sont en partie excessives, notamment s'agissant de la suppression du délai de vingt-quatre heures. Le Gouvernement n'est pas fermé à des évolutions qui permettent de mieux préciser le texte et de prévenir une potentielle surinterprétation des acteurs, mais nous estimons qu'il nous faut conserver un cadre qui fixe le niveau d'ambition pour les réseaux sociaux concernés. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces éléments durant nos débats. Nous avons aussi entendu certaines questions juridiques soulevées notamment par la Commission européenne sur l'articulation de cette proposition de loi avec le cadre réglementaire européen. Il s'agit bien évidemment d'un enjeu important que nous avons pris en compte dès l'origine de ce texte et nous sommes ouverts à affiner encore le dispositif. La commission des lois a entamé cette tâche et je veux saluer l'esprit constructif qui a présidé à ses travaux, sous l'impulsion du rapporteur Frassa. Structurellement, nous nous inscrivons résolument dans une perspective européenne sur ce sujet et, je le dis très clairement, nous soutenons pleinement les pistes esquissées par la Commission européenne que nous avons d'ailleurs appelées de nos voeux depuis le début. Le moment venu, cette régulation devra constituer le cadre de référence.

urgente de la haine en ligne doit être traitée maintenant, et non demain. Un échange récent avec les institutions et les parties prenantes, notamment américaines, de la régulation des contenus me conduit du reste à penser que les travaux menés en France sont observés avec beaucoup d'intérêt à l'étranger, car ils jettent les bases d'une régulation inédite des réseaux sociaux : une régulation agile, capable de s'adapter à des acteurs en perpétuelle transformation, tout en étant ferme pour être véritablement dissuasive. Et les obligations seront d'autant plus fortes qu'elles feront l'objet d'une véritable supervision par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), future autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Je suis convaincu que cette supervision nouvelle des grandes plateformes est la clé d'une régulation beaucoup plus ambitieuse du numérique. Je sais que le Sénat a beaucoup travaillé sur cette question- je pense notamment à l'engagement constant et ancien de la présidente Morin-Desailly et aux initiatives de la commission des affaires économiques -et je ne doute pas que bon nombre d'entre vous seront en phase avec notre volonté de demander plus de comptes aux géants du numérique. Nous avons aujourd'hui la chance de pouvoir poser un jalon historique sur ce sujet essentiel pour l'avenir de nos démocraties et de nourrir les futurs travaux européens qui seront menés sur ces sujets. Mesdames, messieurs les sénateurs, jamais la haine en ligne n'a été aussi visible, destructrice, et jamais le sentiment d'impunité n'a été aussi largement répandu chez nos concitoyens, comme si la vie en ligne autorisait les propos les plus abjects hors le regard de la justice et loin de toute réponse de la société au travers de sanctions. Je n'ignore rien du chemin qu'il nous reste à accomplir pour garantir l'effectivité des mesures que nous prévoyons avec ce texte, mais je connais aussi la détermination en la matière du Président de la République, du Premier ministre et de la garde des sceaux. J'entre dans ce débat avec la volonté de bâtir, avec le Sénat, un texte conforme à l'objectif politique initial et robuste juridiquement. C'est pourquoi j'espère que nous serons en mesure lors des discussions qui s'ouvrent de parfaire les contours de ce cadre équilibré, efficace et ambitieux. Monsieur le Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, en votre nom, j'ai le plaisir de saluer la présence, dans la tribune d'honneur, d'une délégation du Sénat du Royaume hachémite de Jordanie, conduite par son président M. Fayçal Al-Fayez et composée de quatre sénateurs du groupe d'amitié présidé par Mme Haifa Najjar. La délégation est accompagnée par notre collègue Cyril Pellevat, président du groupe d'amitié France-Jordanie. La délégation est en France jusqu'au 19 décembre pour une visite d'étude consacrée notamment aux questions d'éducation et de santé. Elle a été reçue hier en audience par le président Gérard Larcher et s'est entretenue ce matin avec la secrétaire d'État auprès de la ministre des armées. Elle rencontrera en fin de journée les sénateurs de la commission des affaires sociales présidée par notre collègue Alain Milon. Le Sénat français entretient d'excellents rapports de confiance et d'amitié avec le Sénat jordanien. rapports ont vocation à s'intensifier dans le cadre de notre relation bilatérale qui s'est développée autour de deux priorités : la sécurité et l'économie. Mes chers collègues, permettez-moi de souhaiter, en votre nom à tous, à nos homologues du Sénat jordanien la plus cordiale bienvenue, ainsi qu'un excellent et fructueux séjour.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, monsieur le secrétaire le secrétaire d'État, mes chers collègues, la commission des lois a examiné la proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet le 11 décembre dernier. Tous ici sur ces travées nous partageons l'objectif visé : lutter contre la haine en ligne. Pour ce faire, il faut agir d'abord contre ceux qui tiennent des propos haineux et spécialement contre les professionnels de la haine. En la matière, hélas, c'est moins de lois nouvelles que de moyens que nos services ont besoin. agir également sur les intermédiaires techniques, comme le propose ce texte ; cela reste légitime et nécessaire. Certains de ces hébergeurs, dont le modèle économique est fondé sur l'« économie de l'attention », tendent en effet à valoriser la diffusion des contenus les plus clivants, et renforcent la diffusion massive, virale, des messages de haine. Trop longtemps repoussée, leur régulation doit enfin devenir réalité. C'est donc dans un esprit constructif que nous avons abordé l'examen de ce texte au Sénat, en tentant de tenir une délicate ligne de crête entre, d'une part, la protection des victimes de haine et, d'autre part, la protection de la liberté d'expression, telle qu'elle est assurée dans notre pays. quelques regrets sur la méthode, cependant : sur un sujet aussi sensible, alors que la démarche s'inscrit clairement dans le cadre d'un plan gouvernemental global de lutte contre les discriminations, nous regrettons vivement le choix qui a été fait de recourir à une proposition de loi plutôt qu'à un projet de loi, privant de nouveau le Parlement d'une étude d'impact. Nuit aussi à la clarté de nos débats l'existence de trois autres textes adoptés ou en voie de l'être : la directive Services de médias audiovisuels, le règlement européen sur les contenus terroristes et le projet de loi de réforme de l'audiovisuel risquent en effet d'interférer avec certaines dispositions de la présente proposition de loi, voire d'en imposer la réécriture à brève échéance. J'en viens aux modifications adoptées par la commission des lois. Nous avons tout d'abord considéré que l'article 1 comportait un dispositif pénal inabouti et déséquilibré au détriment de la liberté d'expression. En exigeant des opérateurs de plateformes qu'ils apprécient le caractère manifestement illicite des messages haineux signalés dans un délai particulièrement bref, ce dispositif encourage mécaniquement les plateformes à retirer, par excès de prudence, des contenus pourtant licites. En effet, cet exercice de qualification juridique est difficile pour certaines infractions contextuelles, et ce d'autant plus que les plateformes auraient été sous la menace de sanctions pénales lourdes en cas d'erreur. D'autres effets pervers sont également à redouter, comme la multiplication du recours à des filtres automatisés et l'instrumentalisation des signalements par des groupes organisés de pression ou d'influence, à savoir les fameux « raids numériques », contre des contenus licites, mais polémiques. De plus, il pourrait être difficile, voire impossible d'établir la priorité, dans un délai couperet uniforme de vingt-quatre heures, des contenus les plus nocifs qui ont un caractère d'évidence et doivent être retirés encore plus plus rapidement, comme ceux qui touchent au terrorisme et à la pédopornographie, par rapport à d'autres infractions moins graves ou plus longues à qualifier, car elles sont contextuelles. Tout aussi problématiques sont le contournement du juge et l'abandon de la police de la liberté d'expression sur internet aux grandes plateformes étrangères. Le dispositif pénal envisagé semble pour sa part difficilement applicable. Le simple non-retrait suffit-il pour caractériser automatiquement l'infraction, ou est-il nécessaire pour l'autorité chargée de la poursuite de caractériser une absence de diligences normales de l'opérateur, ce qui est beaucoup plus complexe ? À ces difficultés déjà sérieuses s'en est ajoutée une dernière, et non des moindres : la Commission européenne a transmis au Gouvernement des observations longues et très critiques, alertant sur la violation probable de la directive e-commerce et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Selon elle, le texte viole plusieurs principes majeurs du droit européen : le principe du pays d'origine ; la responsabilité atténuée des hébergeurs ; l'interdiction d'instaurer une surveillance généralisée des réseaux. Rappelant l'existence de plusieurs initiatives législatives européennes en cours, la Commission a invité formellement la France à surseoir à l'adoption de ce texte. Faute d'offre alternative crédible, la commission des lois a procédé à la suppression de cette nouvelle sanction pénale inapplicable et contraire au droit européen. Certaines dispositions intéressantes ont, pour leur part, été conservées, améliorées et intégrées au régime général prévu par la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) ajout des injures publiques à caractère discriminatoire et du négationnisme aux contenus devant faire l'objet d'un dispositif technique de notification ; simplification des notifications prévues ; reconnaissance de l'action des associations de protection de l'enfance. Le coeur de ce texte, comme vous l'avez indiqué, monsieur le secrétaire d'État, reste l'imposition d'obligations de moyens sous la supervision d'un régulateur habilité à prononcer des sanctions dissuasives. C'est la solution la plus pertinente pour contraindre les grandes plateformes à une lutte plus efficace contre les discours de haine véhiculés sur les réseaux. Nous l'avons donc approuvée ; nous l'avons même renforcée. La commission des lois a tenu compte des observations de la Commission européenne pour rendre ce dispositif plus respectueux du droit européen en proportionnant les obligations à la charge des plateformes au risque d'atteinte à la dignité humaine et en écartant toute obligation générale de surveillance des réseaux. Pour améliorer la rédaction de certaines des obligations de moyens mises à la charge des plateformes, la commission des lois a l'absence d'information systématique des auteurs de contenus au stade de la simple notification par un tiers, et ce pour éviter les spams et les raids numériques contre les auteurs de contenus licites, mais polémiques. Par ailleurs, à titre exceptionnel, nous avons envisagé la possibilité, dans certains cas, de ne pas informer l'auteur de contenus retirés, notamment pour préserver les enquêtes en cours. Enfin, nous proposons la suppression de l'obligation générale faite aux plateformes d'empêcher la réapparition de tout contenu illicite contraire au droit européen. La commission a aussi approuvé plusieurs clarifications procédurales concernant les pouvoirs de régulation et de sanction attribués au CSA. Je souhaite vous faire part, à cet égard, de ma vive inquiétude, car le régulateur risque de manquer de moyens et de compétences techniques pour expertiser efficacement les plateformes. La commission des lois a, en outre, souhaité compléter le texte pour mieux s'attaquer à la viralité, qui est le coeur du problème de la haine sur internet. Avec la proposition de loi telle qu'elle nous a été transmise par l'Assemblée nationale, une plateforme qui retirerait un contenu haineux vu 8 millions de fois au bout de 23 heures et 59 minutes après une notification respecterait parfaitement l'obligation de résultat que tendait à instaurer l'article 1 ... Selon nous, il faut non pas viser une obligation illusoire de retrait exhaustif de tous les contenus en vingt-quatre heures, mais bien renforcer l'efficacité de la lutte contre les plus viraux et les plus nocifs de ces contenus. Dans ce but, la commission des lois a ajusté la liste des acteurs soumis aux obligations de moyens renforcées de lutte contre les contenus haineux, pour permettre au CSA d'attraire dans le champ de sa régulation des plateformes moins grandes, mais très virales. Elle a aussi encouragé les plateformes, sous le contrôle du CSA, à prévoir des dispositifs techniques de désactivation rapide de certaines fonctionnalités de rediffusion massive des contenus. La commission a également adopté un amendement d'appel visant à mieux associer les régies publicitaires à la lutte contre le financement de sites facilitant la diffusion en ligne des discours de haine par un renforcement des obligations de de transparence à leur charge. Nous y reviendrons. Enfin, comme le recommandait la commission d'enquête du Sénat sur la souveraineté numérique, nous avons souhaité encourager l'interopérabilité pour permettre aux victimes de haine de se réfugier sur d'autres plateformes ayant des politiques de modération différentes, tout en pouvant continuer à échanger avec les contacts qu'elles avaient noués jusqu'ici. Ce travail important

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la commission des affaires économiques s'est saisie pour avis de la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui, car celle-ci modifie la loi pour la confiance dans l'économie numérique de 2004, dite LCEN, dont nous avions été saisis au fond. Même si son objectif relève de la protection des libertés fondamentales, elle affecte donc un secteur qui est aujourd'hui au coeur de la compétence de la commission. Quelques considérations sur la méthode, d'abord. Nous regrettons que, malgré une longue gestation, le Gouvernement ait, de nouveau, choisi une proposition de loi plutôt qu'un projet de loi. voie prive le Parlement d'une étude d'impact qui, en l'espèce, était plus que nécessaire. Nous regrettons également que, malgré nos demandes, nous n'ayons pu prendre connaissance des observations de la Commission européenne que par voie de presse. Tout le monde en disposait, sauf les rapporteurs du Sénat ! Et je passe sur les réponses écrites envoyées moins d'une semaine avant le passage en commission, alors que le questionnaire avait été adressé près de deux mois auparavant J'en viens au fond. Cette proposition de loi s'attaque indéniablement à une question légitime. Si le phénomène est encore peu documenté, chaque utilisateur des réseaux sociaux peut aujourd'hui constater que les propos haineux répréhensibles s'y répandent quotidiennement. Néanmoins, la réponse apportée à cette question est apparue inaboutie. C'est pourquoi nous soutenons le texte issu des délibérations de la commission des lois, qui permet de rendre le dispositif davantage susceptible d'atteindre son objectif, à savoir lutter contre les contenus haineux illicites en ligne, tout en limitant le risque d'atteinte à la liberté d'expression. Les trois commissions saisies ont travaillé en bonne intelligence, avec un seul but : améliorer ce texte pour le rendre plus efficace. La commission des affaires économiques a concentré son analyse sur le dispositif de régulation administrative confié au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). À nos yeux, il est intéressant pour plusieurs raisons. D'abord, il paraît plus efficace et moins attentatoire aux libertés que les dispositions figurant initialement à l'article 1 de la proposition de loi. Il s'agit de prévoir des obligations de moyens, dont la portée est déterminée par un régulateur, lequel est en mesure de sanctionner sévèrement les acteurs qui ne joueraient pas le jeu. La commission des affaires économiques a donc souhaité, en bonne entente avec la commission des lois, renforcer ce mécanisme. C'est pourquoi elle a proposé un amendement qui, dans le droit fil des conclusions de la « mission Facebook permet au CSA d'imposer des obligations à des plateformes de moindre importance, mais sur lesquelles la tenue de propos haineux illicites serait régulièrement constatée. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons souhaité permettre au CSA d'encourager le partage d'informations entre plateformes. Cela nous paraît être le levier essentiel d'une meilleure coopération entre ces dernières et donc d'une lutte plus efficace contre la diffusion de propos punis par la loi. Nous avons également souhaité intégrer au texte un principe de proportionnalité, afin de nous assurer que les obligations de moyens mises à la charge des plateformes seront soutenables par les acteurs économiques, adaptées aux différents modèles que l'on peut trouver sur le marché, et qu'elles prendront en compte la viralité du contenu. Par ailleurs, la commission s'est particulièrement intéressée à ce dispositif en ce qu'il semble poser le premier jalon d'un nouveau modèle de régulation de l'économie numérique. Notre assemblée l'a affirmé à plusieurs reprises, la directive e-commerce n'est pas l'alpha et l'oméga de l'économie numérique. Une régulation intelligente, agile et qui s'applique en priorité aux géants du numérique peut venir la compléter, même si, en l'état du droit européen, la ligne de crête est étroite. La proposition de loi visant à garantir le libre choix du consommateur dans le cyberespace, déposée par notre commission et cosignée par plus de la moitié des membres de notre assemblée, permettra de poursuivre ces travaux tendant à établir un nouveau modèle de régulation de l'économie numérique.

Dans ce contexte, pourquoi sommes-nous collectivement si réticents au dispositif qui nous est soumis ? Au Sénat, nous savons écouter. Or les retours que nous avons des tribunaux, des associations de défense des libertés, des meilleurs spécialistes, bref, de presque tout le monde, sont partagés : il y a ceux qui pensent que

et qui nous conduisent à une approche prudente, circonspecte, de l'article 1 et du retrait en vingt-quatre heures. J'avoue être franchement hostile à l'idée de confier aux Gafam le droit de juger ce qui est licite ou illicite. Ces plateformes qui nous abusent fiscalement, pillent allègrement nos données personnelles pour les revendre et contribuent à manipuler les scrutins se verraient confier un rôle de censeur ... Non seulement elles façonnent toujours plus nos comportements et sont des menaces avérées pour nos démocraties, mais elles pourraient en plus exercer une police de la pensée et de l'expression étant, nous avons la conviction, et de très longue date, au Sénat, qu'il est nécessaire d'avancer sur la régulation du monde numérique. C'est pourquoi nous avons regardé avec attention les autres dispositions du texte, qui précèdent la future loi audiovisuelle. Sur le fond, la commission de la culture s'est saisie des articles 4, relatif à la régulation du CSA, ainsi que 6 et 6 , consacrés à l'éducation au numérique. Sur ce dernier sujet, c'est le Sénat qui a introduit en 2009 la nécessité pour l'école d'informer les élèves sur les risques liés aux usages des services de communication au public en ligne. Depuis, le code de l'éducation s'est enrichi de très nombreuses dispositions relatives à la sensibilisation à propos d'internet, parfois redondantes. Ce qu'il faut, en fait, c'est rapidement donner à l'école les moyens financiers et humains de remplir ce rôle. Cela passe avant tout par la formation initiale et continue des enseignants, comme nous l'avons signalé encore lors des débats sur la loi pour une école de la confiance. En ce qui concerne la régulation, la commission de la culture a adopté plusieurs amendements visant à mieux préciser l'action du CSA. Force est cependant de constater, une nouvelle fois, que nous avons délibérément choisi de remettre une fraction essentielle de notre souveraineté entre les mains d'acteurs mondialisés réticents à toute forme de régulation, et même de discussion, avec des autorités démocratiquement élues, comme l'illustrent jusqu'à la caricature les développements sur les droits voisins des éditeurs et des agences de presse. Ces acteurs ne se contentent pas d'être puissants,

elle a montré que les algorithmes d'une plateforme comme YouTube, c'est-à-dire Google, nourris de milliards de données personnelles collectées sans que l'utilisateur s'en rende compte, produisaient des résultats qui échappent maintenant à notre compréhension, nous rapprochant toujours plus du monstre de Frankenstein. Ils ont donc tendance à proposer des contenus toujours plus odieux, haineux, « de plus en plus hardcore ». Selon cette sociologue, « YouTube est certainement aujourd'hui l'un des plus puissants outils de radicalisation de ce XXI siècle », avec une seule justification : cela fonctionne

comme le propose l'entrepreneur Tariq Krim, le mouvement sur les technologies éthiques. Il s'agit d'un nouveau terrain de croissance industrielle pour l'Europe dans lequel nous aurions tout intérêt à nous investir. Il est soutenu par des entrepreneurs qui réfléchissent à d'autres façons non aliénantes de concevoir la technologie et qui prônent l'arrêt de certaines pratiques

attentistes et inefficaces que nous allons avancer. Cette directive, qui organise notre vie numérique depuis bientôt vingt ans, n'a plus d'autre rôle aujourd'hui que de protéger les monopoles de quelques géants anglo-saxons qui ont actuellement droit de vie et de mort sur nombre de nos entreprises. Il est grand temps de reconnaître qu'elle a échoué à transformer l'Europe en puissance numérique. J'espère que nos discussions de ce jour nous permettront d'y voir plus clair sur les conséquences de ce texte.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues,

Fait rarissime pour une assemblée qui ne refuse jamais de travailler sur un texte, nous avions adopté ces motions, mes chers collègues, à la quasi-unanimité. Nous voulions ainsi alerter le Gouvernement sur la méthode et sur le fond. monsieur le secrétaire d'État, vous aviez choisi la voie d'une proposition de loi inaboutie, dépourvue d'étude d'impact, et discutée dans le cadre de la procédure accélérée.

Il ne les avait pas entendus et je vous montrerai, par l'exemple, que leurs craintes étaient fondées. Aujourd'hui, sans avoir rien appris de ce naufrage, vous récidivez, et vous nous soumettez, dans les mêmes conditions, sans étude d'impact, sans analyse juridique, en recourant à la procédure accélérée, une proposition de loi que vous reprenez à votre compte, alors qu'elle suscite les plus vives réserves de tous les acteurs du numérique, du Conseil national du numérique, du Conseil d'État et même de la Commission européenne, dont vous nous expliquez qu'elle n'est pas défavorable au texte, tout en refusant, en même temps, de nous transmettre son avis. Votre aveuglement vous conduit à la situation cocasse de recevoir des leçons de la République tchèque en matière de défense de la liberté d'expression. Je loue le travail acharné de notre rapporteur, M. Frassa, qui a tenté de rendre conforme un texte de circonstance aux exigences du droit français et européen, et de le transformer en une un peu plus respectueuse des principes constitutionnels relatifs à la liberté d'expression. Cet effort désespéré lui vaudrait sans conteste la médaille de sauvetage, si elle n'était destinée qu'aux seuls Bretons. Néanmoins, plusieurs de vos amendements laissent à penser que sa ténacité restera vaine et que vous imposerez votre rédaction initiale à l'Assemblée nationale. Pour éviter cet échouage, il eût été de bonne méthode de réaliser préalablement un bilan de l'application de la loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information, promulguée voilà bientôt un an. Elle exigeait des opérateurs de plateforme de prendre des mesures pour assurer la transparence de leurs algorithmes, de publier un bilan annuel de leur lutte contre la diffusion des fausses informations, de désigner un représentant légal exerçant les fonctions d'interlocuteur référent sur le territoire français et de communiquer des statistiques sur les résultats des traitements algorithmiques de recommandation et de classement. Le CSA a reçu pour mission de suivre le respect de ces obligations. Un an après le vote de la loi, il a toujours les plus grandes difficultés à obtenir des opérateurs les informations exigées. Cette même loi a créé une action judiciaire en référé pour interrompre rapidement la diffusion d'une information fausse lors d'une campagne électorale. Le Sénat quasi unanime avait exprimé ses plus vives réserves sur l'efficience de ce dispositif. Nous ne disposons pas d'un bilan d'application de cette loi, mais il semblerait que le seul recours dont ait eu à connaître le tribunal de grande instance de Paris soit le mien Je me permets de l'évoquer rapidement dans cette discussion, parce que le jugement rendu, en référé, montre combien la loi est inapplicable et comment les opérateurs peuvent aisément se soustraire à tout contrôle. Le 1 mai dernier, le ministre de l'intérieur a publié sur Tweeter le message suivant : « Ici à la Pitié-Salpêtrière, on a attaqué un hôpital. On a agressé son personnel soignant. Et on a blessé un policier mobilisé pour le protéger ». Plus tard, il reconnaissait lui-même que le mot « attaqué » était inapproprié et le tribunal, dans une litote, a considéré que le message « appara[issait] exagéré en ce qu'il évoqu[ait] le terme d'attaque et de blessure ». il a considéré que chaque électeur avait la possibilité de se faire une opinion plus juste en lisant les articles de la presse écrite et, surtout, qu'il n'est pas possible de déterminer si la promotion de cette information a été assurée par des outils automatisés. Enfin, la société Twitter France a fait valoir son défaut de qualité à agir en précisant que la société Twitter International Company, de droit irlandais, est seule responsable du traitement des données. Aujourd'hui, cette information fausse est toujours disponible et le message a été lu plusieurs milliers de fois. On pressent bien que l'intérêt de la plateforme qui le diffuse tient davantage au débit qu'à la vérité. Elle participe, comme ses homologues, de cette économie de l'attention que vous refusez de réguler, par faiblesse ou connivence. Cette proposition de loi s'intéresse aux conséquences d'un modèle économique que plusieurs d'entre nous, au sein de cette assemblée, vous proposent de juguler, notamment en imposant des dispositifs d'interopérabilité et de transparence des algorithmes. En acceptant les amendements qui les visent, vous manifesteriez, monsieur le secrétaire d'État, votre intention d'agir sur les causes. La parole

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je ne peux, au moment d'examiner cette proposition de loi, m'empêcher d'exprimer ma surprise sur la façon dont la discussion s'engage.

Pour la mettre en oeuvre, nous créons un nouveau délit, placé sous le contrôle du juge. » La raison de cette proposition est assez évidente : la loi pour la confiance dans l'économie numérique, telle qu'elle est rédigée aujourd'hui, se révèle impuissante à enrayer le phénomène de la haine sur internet, qui ne fait que s'amplifier de jour en jour. Je pense que ce constat n'aura échappé à personne ici et que nous sommes tous d'accord. Or, en supprimant la création de ce délit, la commission des lois a retiré de cette proposition de loi ce qui en fait la substance même. Ce qu'il en reste est un texte qui n'a plus grand intérêt. C'est non pas moi qui le dis, mais la Quadrature du Net, et ses membres connaissent le sujet : « Ainsi modifié, le texte n'a presque plus de substance, de sorte qu'il devient inutile de l'adopter.

C'est pourquoi je voterai le texte. » Je cite encore Frédéric Reiss, dans son explication de vote pour le groupe Les Républicains : « J'invite le groupe des Républicains à voter en faveur de cette proposition de loi. » Je cite enfin M. Dunoyer pour le groupe UDI : « Je vais évidemment inciter avec la plus grande conviction les membres du groupe UDI à voter favorablement ce texte.

Vous comprenez mon étonnement ... Pour ma part je suis partisan du texte initial, et je vais essayer, sans me faire d'illusion sur le résultat final, d'en expliquer les Première réflexion : jusqu'à quand les Gafam vont-ils piétiner toutes les règles édictées par nos sociétés démocratiques ? Jamais dans l'histoire des propos publics d'une telle violence, d'une telle infamie, d'une telle obscénité, d'une telle pourriture n'ont été livrés, en toute impunité, à des millions de nos concitoyens. Les écueils des réseaux sociaux sont devenus majeurs,

Deuxième réflexion, qui me paraît devoir aussi faire l'unanimité : la législation actuelle ne permet pas de faire face, puisque le phénomène ne fait qu'empirer. Le temps de la justice ou des autorités administratives n'est pas celui d'internet. Le CSA, l'Arcep (Autorité de régulation des Les seuls qui disposent des énormes moyens humains, algorithmiques et financiers pour régler le problème sont ceux qui l'ont créé. Pour paraphraser un proverbe arabe, celui qui a fait monter l'âne en haut du minaret devra aussi l'en faire redescendre. Troisième réflexion : ce texte reviendrait à une privatisation de la censure, et nous confierions aux plateformes ce qui doit être confié au juge. Eh oui ! Je réponds, d'une part, que c'est bien le juge qui reste l'arbitre en dernière instance, et, d'autre part, que c'est aujourd'hui que la censure existe, et elle est toute-puissante La censure, ce sont les milliers d'internautes qui n'osent plus s'exprimer sur les réseaux sociaux, qui ont résilié leur abonnement pour ne plus s'exposer aux attaques racistes, antisémites, homophobes, sexistes, menées sous forme de raids en bande organisée

Quatrième réflexion : certains objectent que ce texte risque de porter atteinte à la liberté d'expression. Comment peut-on soutenir cette position, alors que le mécanisme va exactement dans le même sens que celui qui s'applique à la presse depuis 1881 ? La loi précise que la presse n'a pas le droit de livrer de contenus haineux ou de diffamer. La presse se conforme depuis toujours à ces principes ; elle contrôle ses contenus et personne n'a jamais dit qu'on lui confiait le rôle du juge. Pourquoi y aurait-il deux poids deux mesures ? L'erreur de raisonnement consiste à distinguer les éditeurs, c'est-à-dire la presse, et les hébergeurs, alors qu'ils ont un point commun : ce sont des diffuseurs. Or c'est la diffusion qui compte en la matière. De ce point de vue, plateformes et presse ont de toute évidence les mêmes responsabilités. La liberté d'expression ne consiste pas à diffuser de la haine, des contenus violents, des appels au meurtre ou au viol ; elle ne consiste pas à empêcher les autres de s'exprimer par du harcèlement, des attaques massives ou des menaces. En confondant ces délits avec la liberté d'expression, ce sont, non pas les victimes, mais les agresseurs On nous dit, enfin, que la Commission européenne est hostile à ce texte. Elle est surtout hostile à ce qu'il révèle : elle n'a rien fait depuis des années ! La directive e-commerce date de 2000, à un moment où aucune des plateformes actuelles n'existait, ou presque. La présente proposition de loi va, évidemment, bien au-delà de cette directive, qui est d'un laxisme inimaginable, comme de nombreux textes européens dans ce domaine, gangrénés par les millions de dollars du lobbying des Gafam à Bruxelles. Ce n'est que lorsque certains pays ont commencé à légiférer

et, comme d'habitude, elle nous dit : « c'est notre affaire, pas la vôtre ! » Je pense, pour ma part, que l'inaction passée n'est pas un gage d'efficacité future et que nous aurions tout à gagner à bousculer un peu la Commission européenne, plutôt que d'attendre qu'elle sorte de sa torpeur.

nombre de nos concitoyens, avons été les témoins, souvent impuissants, de propos haineux sur internet. Il a même pu arriver que nous en soyons les cibles. Il n'est donc pas nécessaire de dresser un florilège des expressions odieuses, souvent anonymes, qui sont apparues progressivement avec le développement de cet outil de communication qu'est internet. Chacun sait ce qu'est l'expression de la haine raciste, antisémite, négationniste, l'apologie du terrorisme ou des crimes contre l'humanité, l'incitation à la haine en raison d'un handicap, d'une appartenance réelle ou supposée à une orientation sexuelle, d'une orientation politique, d'une croyance religieuse.

partagent les objectifs visés en l'espèce- c'est d'ailleurs, je crois, notre cas à tous. Force est de constater que le droit en vigueur, qu'il s'agisse du droit français ou du droit européen, ne nous permet pas de lutter efficacement contre l'expression de la haine en ligne. Nous sommes donc convaincus de la nécessité de renforcer l'arsenal législatif dédié à cette lutte, pour l'adapter aux nouveaux supports que cette haine emprunte pour proliférer. Oui, il faut trouver un moyen pour qu'un contenu haineux puisse être signalé, supprimé, et sa viralité anéantie. Mais, monsieur Malhuret, pas au prix de l'atteinte à une liberté constitutionnelle J'ai déjà exprimé notre inquiétude sur les moyens potentiellement attentatoires aux libertés mis en oeuvre au motif de défendre la sécurité et l'ordre public. Malheureusement, le constat s'impose à tous : depuis deux ans, l'actuelle majorité s'est fréquemment heurtée à cet écueil au prétexte de l'efficacité et a souvent consenti à ébrécher les libertés publiques. Ne commettons pas, de nouveau, cette erreur morale

Or c'est à l'aune d'un postulat de départ plaçant la liberté au second plan, derrière la recherche de l'efficacité, que certaines dispositions de ce texte, pourtant centrales, s'avèrent problématiques et que certains manques se révèlent préoccupants. En la matière, la recherche de l'efficacité revêt la forme de la prédominance donnée au contrôle privé, par les plateformes, au détriment du juge judiciaire, seul compétent, selon moi, en matière de limitation de la liberté d'expression.

La Commission européenne a pour sa part émis des observations très préoccupantes, dont la prise en compte pourrait justifier le rejet de toute demande de condamnation d'une plateforme par un juge français. Nous avons donc le devoir d'adapter notre droit aux évolutions du temps, mais nous devons absolument en préserver les principes fondamentaux. C'est l'objectif visé par mon groupe. Quelles sont nos préoccupations ? En premier lieu, les auteurs du texte n'ont pas jugé nécessaire de distinguer les organes de presse parmi les auteurs de contenus. Ce serait un oubli lourd de conséquences, si la future loi restait en l'état en ce domaine. Il est donc impératif que le Sénat défende la liberté de la presse en l'excluant du champ de la loi. Nous y reviendrons. second lieu, un certain nombre de garde-fous doivent être mis en place. D'abord, il y a le fameux délai de vingt-quatre heures laissé à un opérateur pour déterminer si le contenu notifié est haineux ou non, et s'il doit être retiré ou non. Cette mesure a été vivement critiquée, non sans raison. Ce délai conduit à s'interroger effectivement sur les décisions nécessairement radicales qui pourraient être prises par les plateformes numériques,

Pour autant, il est primordial que nos travaux confèrent à ce texte les moyens de lutter efficacement contre la haine en ligne. Le groupe socialiste avance un certain nombre de propositions pour dépasser cette problématique, en renforçant le rôle du juge.

une obligation de retrait ou de blocage en vingt-quatre heures à titre provisoire d'un contenu haineux manifestement illicite notifié, jusqu'à sa validation par le tribunal de grande instance statuant en référé. Nous pensons enfin qu'il convient d'aller plus loin encore dans le rôle conféré au CSA dans le dispositif. En organisant sous son autorité la coopération et le partage transparent d'informations entre les plateformes,

Le CSA doit également assurer son rôle d'autorité de régulation et de contrôle pour ce qui concerne les algorithmes utilisés par les plateformes en matière de suggestion et d'accès aux utilisateurs de certains contenus. Les moyens doivent lui être donnés d'assurer ces missions et d'en garantir la transparence. À défaut, nous serons pieds et poings liés face aux plateformes, qui pourront, grâce à des algorithmes que nous ne connaîtrons pas par hypothèse, censurer toute une série de contenus. D'autres points méritent amélioration. Ils seront évoqués par mon collègue David Assouline dans quelques instants. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le groupe socialiste aborde l'examen de ce texte avec un esprit de responsabilité. C'est le sens des amendements que nous proposerons : il s'agit bien de répondre aux deux exigences d'efficacité et de justice, à travers une lutte contre la haine sur internet

la ministre, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, depuis de nombreuses années, nous faisons face à une explosion du racisme et de l'antisémitisme en ligne. Aussi, l'objectif de cette proposition de loi est partagé sur l'ensemble de nos travées. Il était important d'agir face au déferlement de haine Cette avalanche de haine est d'autant plus méprisable qu'elle se fait souvent sous le sceau d'un relatif anonymat, qu'une enquête approfondie finit bien souvent par trahir. Pour en venir à la proposition de loi, la version issue des travaux de l'Assemblée nationale posait à mon sens un certain nombre de difficultés. La création d'un délit de non-retrait des contenus odieux dans un délai de vingt-quatre heures, à l'article 1, constituait la principale de ces difficultés. L'instauration d'un tel délit aurait comme première conséquence de confier la censure sur le web à des géants de l'internet mettant déjà à mal la souveraineté des États. Ces géants auraient été d'autant plus confortés que le texte initial prévoyait de sanctionner en fonction du nombre de connexions, lequel ne détermine en rien les moyens d'une plateforme. C'est simple, on aurait sanctionné de la même manière Facebook, ayant une véritable portée commerciale, et Wikipédia, qui n'a aucune vocation commerciale et dont la communauté régule déjà les contenus.

problème soulevé par ce délai, enfin, est qu'il mettait tous les propos haineux au même niveau, empêchant ainsi toute possibilité de s'attaquer, d'abord, aux atteintes jugées les plus lourdes. Tous ces éléments rendaient cette disposition inapplicable. C'est pourquoi je me réjouis de sa suppression par le rapporteur. S'agissant des opérateurs concernés, je salue l'exclusion des moteurs de recherche du champ d'application de la loi. La possibilité que des sites de plus petite ampleur puissent être sanctionnés grâce au critère de viralité mis en place est intéressante, mais les critères de choix énoncés sont trop vagues et laissent une trop grande place à la libre appréciation du CSA. La proportionnalité des moyens selon la taille des plateformes est également une bonne réponse apportée aux critiques formulées par la commission sur la nécessaire hétérogénéité des modèles de plateformes. Quant aux pouvoirs de régulation et de sanction attribués au CSA, le rôle du Conseil relatif à la diffusion de lignes directrices et de bonnes pratiques doit être central pour permettre une mise en oeuvre la plus simple possible de la future loi. J'en reviens à la lutte contre la viralité. Là encore, le CSA aura un rôle majeur à jouer. Les prérogatives qui lui ont été données pour désactiver de manière rapide certains canaux de rediffusion vont aussi dans le bon sens, mais cette montée en gamme pose un problème : celui du financement. Une fois de plus, on va faire supporter davantage de prérogatives et d'obligations à un organisme sans augmenter considérablement ses moyens. Donnons au CSA les moyens de ses ambitions ! Le même raisonnement s'applique pour l'éducation nationale : on lui assigne aujourd'hui des nouvelles missions de sensibilisation auprès des élèves, mais, sans moyens importants, la promesse est vaine. Dans la lutte contre la haine en ligne, le principal défi sera celui de l'interopérabilité des grandes plateformes. Derrière ce mot complexe, se cache simplement la possibilité de mise en place de protocoles communs, permettant la communication entre logiciels. L'objectif à terme est d'arriver à faire sortir certains

utilisateurs de certains usages nocifs des réseaux sociaux et de les éloigner de pratiques souvent peu respectueuses de la vie privée et de la protection des données personnelles. Dans ce domaine, le texte permet quelques avancées, hélas insuffisantes pour bouleverser les équilibres établis par les géants du net.

internet peut être un formidable outil de partage et d'expression, un espace de liberté qu'il nous faut impérativement préserver. Néanmoins, il arrive de plus en plus souvent que son utilisation soit dévoyée. Associé au sentiment d'impunité lié à l'anonymat ou à la virtualité, il est aujourd'hui devenu le lieu privilégié de la prolifération et de la propagation de contenus violents, haineux, ou encore de fausses informations et autres théories du complot. Nous en sommes quotidiennement témoins, si ce n'est victimes. Ces comportements intolérables ont des conséquences parfois dramatiques, devant lesquelles le législateur ne saurait rester silencieux. Il s'agit d'un constat unanimement partagé sur toutes les travées de cette assemblée il est de notre responsabilité d'agir, tout en trouvant un équilibre entre modération des contenus et respect de la liberté d'expression. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui, portée par la députée Laetitia Avia, dont je souhaite saluer le travail considérable, s'attaque à cette tâche difficile. Issue d'un rapport remis en septembre 2018 au Premier ministre par son auteure elle-même, Karim Amellal et Gil Taïeb, elle a pour ambition de renforcer la pression sur les plateformes numériques, en les soumettant à des sanctions pénales si elles ne retirent pas en vingt-quatre heures les contenus et met en place une régulation administrative ambitieuse de ces grandes plateformes placée sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce texte facilite également l'organisation de la réponse judiciaire par la spécialisation d'un parquet et d'une juridiction en matière de lutte contre la haine en ligne. Enfin, il promeut certaines actions de prévention en milieu scolaire. La révolution numérique a grandement modifié les comportements, notamment chez les plus jeunes, qui sont les premiers utilisateurs d'internet. Ce fait justifie que l'on mise sur la prévention, la sensibilisation, l'éducation et la responsabilisation au numérique. Inspirée du précédent allemand, entré en vigueur le 1 janvier 2018, la proposition de loi s'efforçait, me semble-t-il, d'en éviter les écueils. Depuis son dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale, le 20 mars 2019, ce texte a beaucoup évolué, pour tenir compte, notamment, de l'avis du Conseil d'État en date du 16 mai 2019.

La commission des lois du Sénat, par la voix de son rapporteur, M. Christophe-André Frassa, dont je salue la qualité du travail, a choisi de supprimer ce nouveau délit dit de « non-retrait que nous proposions au contraire de préciser, au motif que celui-ci inciterait les plateformes à retirer des contenus licites au moindre doute, par excès de prudence et peur d'une éventuelle sanction. Ce sont des arguments que nous comprenons, même si nous pensons que le texte était parvenu à un équilibre en laissant à la justice le soin de trancher, en cas de contestation, sur le respect de ces obligations de retrait ou, au contraire, en cas de retrait abusif. Nous avons par ailleurs déposé un certain nombre d'amendements, qui ont été adoptés en commission. Je pense à celui qui vise à mieux associer les régies publicitaires à la lutte contre le financement des sites facilitant la diffusion en ligne des discours de haine, en renforçant les obligations de transparence qui leur incombent. Je pense aussi à la suppression de l'obligation mise à la charge des plateformes d'empêcher, de façon générale et indiscriminée, la réapparition de contenus haineux illicites déjà retirés. Cette procédure de était manifestement de était manifestement contraire au droit de l'Union européenne, la directive e-commerce interdisant toute forme de surveillance généralisée des réseaux. Je pense enfin à l'amendement tendant à préciser que le CSA prend en compte l'hétérogénéité des modèles de plateforme dans l'appréciation des moyens mis en oeuvre.

nous sommes tous d'accord pour reconnaître que les grandes plateformes doivent être davantage responsabilisées, afin qu'elles participent bien plus qu'aujourd'hui à la lutte contre la propagation des discours de haine en ligne. Notre législation actuelle, la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, qui se contente d'imposer aux hébergeurs d'agir « promptement » pour retirer les contenus manifestement illicites qui leur sont signalés, n'est plus adaptée. Nous pouvons nous féliciter qu'une action ait été entreprise à l'échelon national, même s'il nous paraît évident qu'une législation harmonisée au plan européen permettrait une réponse plus efficace dans cette lutte contre la haine en ligne. Pour toutes ces raisons, et compte tenu du fait que le texte a été amputé de l'une de ses dispositions principales, le groupe La République En Marche s'abstiendra. La haine en ligne évolue sans cesse, au gré des progrès techniques. Le dispositif mis en place devra faire ses preuves, et il y a fort à parier que nous serons contraints, tant les changements sur internet sont rapides, de remettre l'ouvrage sur le métier et de faire de nouveau évoluer notre loi.

du premier point, qui est de savoir si notre société doit s'armer pour lutter contre les contenus haineux sur internet, la réponse est bien sûr

pas de dispositions pénales, ce qui explique pourquoi la Commission européenne a pris une autre position à son sujet, et le législateur allemand a fixé les éléments de l'obligation de moyens, bien qu'il y ait aussi un régulateur. En conclusion,

sur lesquelles nous siégions, nous aimerions pouvoir trouver une juste réponse, c'est-à-dire opposer la loi de la République à la loi de la jungle digitale.

que la commission des lois a profondément et heureusement modifié : il s'agit de donner un pouvoir de suppression de contenus à ces plateformes internationales.

dispositifs plus opérationnels, tout en protégeant nos libertés en termes de viralité, de célérité et d'interopérabilité pour que ceux et celles qui pourraient être concernés par cette haine- il faut bien sûr la dénoncer et la condamner -puissent se réfugier sur d'autres plateformes.

cette faculté de censure serait concédée non pas à des hommes ou à des femmes, mais à des robots, à des algorithmes dont nous ne connaîtrons jamais les codes sources, mes chers collègues. Voilà le problème ! Ce n'est pas une société de vigilance qu'on nous propose, c'est une société d'une surveillance généralisée. Nous ne le voulons pas.

Le risque de sur-blocage préventif des propos qui pourraient être tenus a déjà été dénoncé. Pour certains, c'est tout à fait louable, car cela permettrait à internet de devenir le lieu d'une aimable conversation civique. civique. Je crains que nous ne puissions d'ores et déjà dessiner les contours de cette aimable conversation civique. En effet, vous le savez sans doute, l'une des plateformes les plus connues proscrit toutes les images de nudité

qui expurgent soigneusement tous les ouvrages, tous les manuscrits, de tous les éléments qui pourraient blesser des groupes d'intérêt, des communautés particulières, si bien que les ouvrages qui en sortent ont à peu près la densité de. Par ailleurs, depuis le 1

que douze victimes sont tombées sous les balles de terroristes islamistes ... Derrière cette volonté tout à fait louable de mettre fin à ces flots insensés de violence qui déferlent en permanence sur la toile se cache la liberté d'expression. C'est une liberté constitutionnelle, c'est l'essence même de notre démocratie, au point que tous les régimes totalitaires cherchent à empêcher leurs citoyens d'aller sur internet.

Je soutiens bien évidemment cette position, car je ne voudrais pas, pour citer un auteur français, pouvoir dire comme Le Figaro de Beaumarchais : « Pourvu que je ne parle en mes écrits ni de l'autorité, ni du culte, ni de la politique, ni de la morale, ni des gens en place [ ...], ni de personne qui tienne à quelque chose, je puis tout imprimer librement sous l'inspection de deux ou trois censeurs. » La parole est à M.

la possible atteinte à la liberté de la presse, qui est constitutive de la liberté d'expression dans notre pays.

Ne pas inscrire ce cadre dans la loi ferait prendre le risque de laisser cette liberté passer sous le joug des plateformes. Or, nous le savons, malgré toutes nos précautions, le risque de voir des algorithmes ne pas tenir compte du contexte et censurer des articles de presse La presse en ligne est d'autant plus sensible qu'elle offre des espaces de contributions qui pourraient apparaître comme des opinions, mais sont pourtant déjà modérées par des éditeurs agréés et couvertes par la loi de 1881.

sous peine de sanction pénale. Nous n'introduisons pas de sanction pénale. Nous multiplions l'amende par quatre et nous changeons « promptement » et

En attendant, prenons un certain nombre de dispositions en France pour protéger les Français. Lorsque les dispositions européennes seront adoptées, elles auront vocation à s'appliquer.

et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. Les atteintes portées à cette liberté doivent donc être nécessaires, adaptées et proportionnées ». Il s'agit d'une exigence extrêmement puissante qui trouve ses racines au fondement même de la démocratie. Nous devons donc assurer cet équilibre.

même si l'existence de règles déontologiques limite, en principe, le risque de diffusion de contenus haineux par les entreprises de presse. Il serait donc, me semble-t-il, difficilement justifiable de traiter différemment un contenu haineux selon qu'il a été ou

À chaque type d'événement sa loi, même si les textes en vigueur permettent d'y répondre ! Dans le cas présent, il y a la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, qu'il suffisait d'adapter. Il y a surtout l'inoxydable loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Les associations militantes l'utilisent sans modération devant la justice,

texte énumère les traites des noirs en oubliant celles vers les pays arabo-musulmans, pourtant plus longues et plus importantes en nombre que la traite transatlantique. Mais, dans notre cas, le problème de fond, c'est que le mot « haine » ne signifie plus grand-chose à force d'être galvaudé ! Aussi en arrive-t-on à énumérer des haines à tour de bras,

texte sera, dans son application, focalisé sur les haines contre les minorités ethniques, religieuses et sexuelles, mais négligera à coup sûr les haines contre la majorité et la haine ordinaire entre les individus,

On peut soumettre les algorithmes à nos valeurs humanistes et libérales, au sens philosophique du mot : donnons-nous les moyens humains et financiers d'y parvenir. Monsieur le secrétaire d'État, vous l'avez annoncé devant notre commission d'enquête : vous allez consacrer des moyens importants au recrutement de scientifiques de très haut niveau,

l'interdiction de vendre du tabac en ligne ne requiert aucune appréciation de licéité de la part des opérateurs de plateforme en ligne. Le retrait de ce type de contenus ne risque donc de porter atteinte ni à la liberté d'expression ni au commerce en ligne licite.

s'agissant des injures discriminatoires, le dispositif vise des propos pour lesquels aucune contextualisation n'est nécessaire pour caractériser l'infraction. Le non-respect de l'obligation de retrait constituera un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 250 000 euros d'amende. Les personnes morales, principalement visées par ce délit, encourront une amende de 1,25 million d'euros et les peines complémentaires d'affichage et de diffusion de la décision de condamnation et d'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. Contrairement à ce qui a été précédemment affirmé, ce dispositif est conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

qui est des contenus visés, le Gouvernement propose d'exclure du dispositif quelques infractions qui ne peuvent être caractérisées à raison d'un contenu, comme les infractions de proxénétisme. Par

je reconnais bien volontiers l'importance de protéger l'activité de nos buralistes ; mais j'ai quelques difficultés à mettre sur le même plan, au sein d'une énumération, je le répète, déjà fort longue, l'apologie des crimes contre l'humanité et la vente de cigarettes sur internet

notre commission, insatisfaisante. Il s'agit toujours d'une obligation de résultat, et les retraits doivent être exhaustifs, c'est-à-dire que tous les contenus manifestement haineux sont concernés, de surcroît dans un délai couperet de vingt-quatre heures, sans aucune souplesse en fonction des circonstances ou du type de contenus. Ainsi, le dispositif envisagé reste déséquilibré au détriment de la liberté d'expression. Il ne manquera pas d'entraîner de nombreux effets pervers : sur-censure, c'est-à-dire blocage par précaution de propos pourtant licites, recours encore plus massif à des filtres automatisés,

problème d'imputabilité se pose tout d'abord, s'agissant des personnes physiques- qui, du modérateur sous-traitant indien ou du dirigeant américain, sera poursuivi ? -et, surtout, des personnes morales- comment qualifier l'intention pénale des organes dirigeants des hébergeurs concernés, domiciliés à l'étranger, dont il faut démontrer la complicité ? Un autre problème se pose, de caractérisation de l'intentionnalité : le simple non-retrait suffira-t-il,

les infractions de presse, qui dépendent beaucoup de leur contexte- ironie, provocation ... Enfin, je répète que, selon la Commission européenne, ce dispositif viole plusieurs principes majeurs du droit européen : la

Mme de la Gontrie vise à réaffirmer le rôle de l'autorité judiciaire pour apprécier le caractère illicite des contenus haineux. Il s'agit d'introduire une sorte de référé-confirmation : les contenus haineux notifiés devraient être retirés temporairement par tout intermédiaire technique, lequel ferait valider sa décision par le juge des référés.

nous nous rejoignons : la faculté donnée à chacun de communiquer et de s'exprimer librement en partageant des contenus sur internet suppose un équilibre délicat entre la liberté reconnue aux personnes et la protection des droits d'autrui ; en France, traditionnellement, l'une des garanties essentielles pour assurer cet équilibre repose sur l'intervention de l'autorité judiciaire.

Cette mesure conduirait immanquablement à engorger nos juridictions au-delà du raisonnable. En outre, la procédure resterait à l'initiative des seuls intermédiaires techniques ; elle représenterait donc une charge importante pour eux.

; mais il me semble qu'il serait extrêmement difficile de rendre automatique la saisine d'un juge des référés qui devrait se prononcer dans un délai très court. Au reste, je crois que votre souhait est satisfait, puisque les auteurs disposent déjà de la possibilité de saisir un juge des référés

votre amendement. Par ailleurs, l'article 3 de la proposition de loi met à la charge des opérateurs des obligations d'information sur l'existence de dispositifs de recours, à destination non seulement des victimes des contenus, mais également des auteurs qui pourraient faire l'objet de la

suivant la procédure de signalement mise en place par la loi de 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, il est remplacé par un message mentionnant la suppression. Nous considérons que cette disposition, si elle est bien utile, n'est pas suffisante

Claude Malhuret. Selon la rédaction actuelle du texte, les contenus ayant fait l'objet d'une notification au sens de la loi pour la confiance dans l'économie numérique et ayant été rendus inaccessibles par un hébergeur

d'apprécier et de qualifier les faits et les circonstances. La simple faculté de conservation ne garantit pas que toutes les infractions pourront être poursuivies. C'est pourquoi le présent amendement vise à rendre la conservation obligatoire pour les besoins de la justice, afin que les infractions constituées puissent être effectivement poursuivies et sanctionnées. La rédaction initiale de mon amendement visait les contenus rendus inaccessibles, sans autre précision.

il me semble important que tous les contenus retirés par les plateformes soient conservés par elles, non seulement les contenus illicites, mais également ceux qui ne le sont pas, pour que la justice puisse sanctionner les retraits abusifs. Si un hébergeur est contraint,

étant donné la surcharge des tribunaux ; il faut considérer en plus les délais de recours. Il est donc indispensable que les contenus haineux soient conservés plus longtemps.

ont un objet commun : instaurer une obligation de conservation des contenus illicites retirés par les hébergeurs, afin de faciliter d'éventuelles poursuites ultérieures. Il s'agit de réaliser un équilibre délicat entre la facilitation des enquêtes et les contraintes imposées aux hébergeurs. D'un côté, il est vrai que l'un des obstacles aux poursuites est trop souvent la disparition des preuves. Lors de l'audition des représentants de la plateforme Pharos, certains enquêteurs ont déploré que les plateformes soient parfois, paradoxalement,

être mentionnée dans la loi. M. Malhuret, lui, renvoie ces modalités à un décret en Conseil d'État- ce qui me semble préférable -pris après avis de la CNIL- ce qui me semble indispensable. Pour ces raisons, j'émets un avis favorable sur l'amendement n° 12 rectifié , et je demande le retrait

hasardeux sur le point de départ de la computation du délai, de la prescription, de l'infraction, etc. Étant favorable à la clarté, je suis, comme le rapporteur, plutôt défavorable au sous-amendement du Gouvernement.

de retrait en une heure des contenus à caractère terroriste ou pédopornographique. Il n'est donc pas du tout de pure coordination, comme peut le laisser penser une lecture rapide de son objet. s'inspire d'un règlement européen actuellement en cours de négociation et tend à créer une obligation de retrait en une heure des contenus à caractère terroriste ou pédopornographique notifiés par l'administration aux hébergeurs et aux éditeurs. Sa méconnaissance serait pénalement sanctionnée, à raison d'un an de prison et de 250 000 euros d'amende portés au quintuple pour les personnes morales. Avant d'aborder le fond, permettez-moi de protester solennellement sur la méthode du Gouvernement qui nous fait ce que je pourrais appeler une mauvaise manière. Déposer un amendement aussi important en le présentant comme un amendement la veille de l'examen en séance auprès de la deuxième assemblée saisie, sans étude d'impact, sans que nous ayons pu interroger précisément les services concernés sur ce qui justifie une telle extension de leurs pouvoirs, n'est pas très respectueux de la qualité du travail parlementaire. La gravité d'un tel tel sujet mériterait une analyse poussée, que les délais contraints ne vont pas permettre de mener de façon totalement satisfaisante. J'en viens au fond. En l'état du droit, si l'éditeur ou l'hébergeur ne répondent pas heures aux demandes de l'administration, celle-ci peut enjoindre les fournisseurs d'accès de procéder au blocage administratif des sites terroristes ou pédopornographiques. Ce blocage échappe au contrôle préalable d'un juge. Le Conseil constitutionnel a admis cette exception en raison du caractère d'évidence et d'extrême gravité des infractions poursuivies. En outre, une personnalité qualifiée indépendante s'assure de la justification de la mesure. L'amendement n° 53 vise à faire peser la charge du blocage administratif directement sur les éditeurs et les hébergeurs, blocage

dont cette mesure s'inspire fait encore l'objet de vifs débats, la commission des lois a souhaité attendre son adoption avant d'envisager de modifier aussi hâtivement notre droit. Le blocage administratif actuel fonctionne bien, et le Gouvernement ne justifie pas dans l'exposé des motifs de la nécessité de légiférer ainsi en urgence. Tous les hébergeurs ne seraient pas matériellement en mesure de répondre en une heure ; seules les grandes plateformes en ont les moyens. Le dispositif proposé est enfin très déséquilibré, puisqu'il ne prévoit aucune des principales garanties envisagées par le projet de règlement européen. Il y a des cas de force majeure ou d'impossibilité technique insurmontable : il faudrait donc prévoir des cas d'exonération de responsabilité. Il y a aussi des cas d'erreur de l'administration : il faudrait donc prévoir de préserver les contenus retirés pour les rétablir à la demande de la personnalité qualifiée ou du juge. Dans ces conditions, je ne peux émettre qu'un avis défavorable

En effet, celle-ci est tenue de le protéger contre les atteintes volontaires à son intégrité, les violences, les agissements consécutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. amendement, notre collègue Jean-Pierre Grand propose d'élargir le bénéfice de cette nécessaire protection des agents publics lorsqu'ils sont victimes de la diffusion de contenus haineux sur internet.

Or, à ce jour, aucun d'entre eux n'a bénéficié de mesures de protection de la part de leur autorité hiérarchique, les laissant ainsi seuls face à des contenus toujours en ligne. Quel est l'avis de la

aux victimes de contenus haineux pour effectuer, à leur place et en leur nom, la notification auprès des hébergeurs des infractions dont ils sont victimes ou témoins sur internet. Cette disposition viendrait donc en complément d'autres dispositions introduites dans la proposition de loi pour faciliter leur action et renforcer leur mission. Ainsi, l'obligation de désigner un représentant légal est bienvenue, car, lorsque des associations souhaitent signaler un message litigieux, elles peinent parfois à identifier un interlocuteur français. Nous souhaitons par cet amendement qu'elles puissent intervenir facilement dans la chaîne de procédure de signalement des contenus illégaux. Il serait même opportun de créer un label officiel de signaleurs de confiance,

plus d'objet. En effet, le nouveau délit de non-retrait de contentieux ayant été supprimé, il n'y a plus de sens à donner intérêt à agir aux associations en vue d'exercer spécifiquement les droits de la partie civile pour poursuivre ce délit. Je tiens que demeure bien entendu inchangée la capacité des associations spécialisées à poursuivre les délits que constituent certains messages haineux eux-mêmes- provocation à la haine raciale, injures sexistes, etc.

travaillent dans le secteur de la protection de l'enfance et ont acquis une sérieuse expérience. Il serait dommageable de leur refuser le droit d'agir car leurs statuts n'auraient pas prévu la mention de leur protection « dans le cadre de leur usage des plateformes en ligne ». Le présent amendement a donc pour objet d'assurer une meilleure protection des mineurs. Quel est l'avis de la Cet amendement proposé par Mme Goulet vise à élargir aux associations exerçant dans le secteur de la protection de l'enfance la possibilité de notifier des contenus haineux à la demande d'un mineur. Ne serait plus exigée la condition spécifique d'une action de protection dans le cadre de leur usage des plateformes en ligne. L'adoption de l'amendement